prétendue irresponsabilité des patients ou par un manque de considération à l'égard des soignants, plusieurs études démontrent que la majorité des patients absentéistes sont en situation de précarité

Aussi nous opposons-nous à cet article, qui stigmatise des patients avant tout des victimes des dysfonctionnements de notre système de santé, à commencer par l'ubérisation

Pénaliser, pour autant que cela soit possible, sans analyser le problème risque de se révéler une solution de faible efficacité. En revanche, cette mesure va précariser des patients qui sont déjà socialement En effet, les études indiquent que les patients en tiers payant social manquent plus fréquemment leurs rendez-vous. Dans sa thèse, le docteur Francis Gatier démontre que « les absences aux rendez-vous des patients précaires surviennent dans le contexte d'un quotidien difficile où la santé n'est pas forcément une priorité ». Parmi les

ou auxquels les patients ne se présentent jamais réduisent inutilement la file active des professionnels de santé. Le dispositif que nous proposons vise à responsabiliser les patients pour dissuader les comportements non vertueux, et non pas à pénaliser sans discernement les patients.

de résoudre l'équation suivante : responsabiliser les patients sans mettre en péril leur accès aux soins et regagner du temps médical sans créer de risques de fraude sociale.

si seuls les syndicats de médecins nous ont alertés lors de leurs auditions sur les difficultés auxquelles ils font face en raison des rendez-vous non honorés, il apparaît nécessaire d'étendre à tous les professionnels de santé le dispositif de l'article 3 . L'amendement vise en outre à corriger une erreur rédactionnelle.

Depuis la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, les assistants dentaires peuvent assister le chirurgien-dentiste ou le médecin intervenant en chirurgie dentaire et contribuer aux activités de prévention et d'éducation à la

prophylactique et orthodontique, ainsi qu'à des soins post-chirurgicaux. Selon l'ordre des chirurgiens-dentistes, la formation nécessaire pour acquérir de telles compétences pourrait se dérouler en deux ans, dans le cadre d'une formation continue. La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle des cabinets dentaires et le ministère de la santé et de la prévention travaillent à la maquette de cette formation diplômante. Mme la rapporteure a conditionné l'accomplissement des nouvelles missions à une formation spécifique.

prohibitifs pour une qualité peut-être incertaine. Renforcer l'attractivité des métiers passe, selon nous, par une revalorisation du rôle des universités, en l'occurrence des facultés de chirurgie dentaire. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement

de discussions entre la branche professionnelle et le ministère. M. le ministre pourra confirmer l'état des échanges, mais la formation pourrait prendre en compte l'expérience des assistants dentaires, se dérouler en alternance et ne pas être nécessairement

consolider la formation des futurs assistants dentaires. Ceux qui sont en exercice suivent une formation dispensée par des centres de formation agréés par la branche.

La responsabilité est pour nous essentielle, car elle est la seule à permettre qu'une phrase figurant dans un texte voté devienne une réalité dans nos territoires. La mention « collective » l'est tout autant, car c'est uniquement en collaborant avec les professionnels de santé

par les agences régionales de santé. Encore une fois, la collaboration doit être au coeur du modèle que nous proposons, au plus près des territoires, en prenant en compte l'avis de ceux qui les connaissent le mieux et surtout de ceux qui, demain, devront être les acteurs centraux de la permanence des soins.

des professionnels en matière de permanence des soins, lesquelles ont été supprimées par la commission. En effet, ces dispositions ne reviennent pas sur le principe du volontariat et inquiètent inutilement les professionnels. C'est la raison pour laquelle la commission a choisi de les supprimer, tout en laissant subsister les dispositions qui permettent aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes et aux infirmiers de participer à la permanence des soins dans leur domaine de compétence respectif. La commission a donc émis un avis défavorable sur l'amendement n°

Les CPTS participent déjà à la mise en oeuvre de la permanence des soins, quand elles existent sur le territoire. Je rappelle, par ailleurs, que la permanence des soins est assurée dans 96 % des territoires les week-ends et dans 95 % d'entre eux en soirée.

de vingt-trois heures. Quel est l'avis de la commission ? Les modalités d'organisation de la permanence des soins sont définies localement par les agences régionales de santé, qui établissent un cahier des charges régional tenant compte des besoins de soins non programmés. Si la permanence des soins ambulatoires est très largement assurée en soirée et le week-end, le niveau de couverture est en revanche d'ores et déjà beaucoup plus faible en nuit profonde : le Conseil national de l'ordre des médecins fait état de 77 % de zones blanches. La commission préfère laisser aux agences régionales de santé le soin de définir les modalités d'organisation les mieux adaptées aux besoins de chaque territoire. L'expression « a vocation à » est déjà utilisée dans le code de la santé publique. Elle ne modifie en

La voie du conventionnement sélectif permettrait de réguler l'installation des médecins. Des précédents existent, qui ont montré leur efficacité. Des professions médicales ou paramédicales sont déjà soumises à une obligation d'installation dans des zones insuffisamment desservies, par le biais du conventionnement, la convention nationale de la profession avec l'assurance maladie est habilitée à subordonner le conventionnement d'un professionnel à son installation dans une zone tendue. Par ailleurs, la régulation, qui s'oppose moins frontalement à la liberté d'installation des médecins, est présentée comme une troisième voie équilibrée entre l'incitation et la coercition. Le conventionnement d'un médecin à l'assurance maladie ne serait ainsi autorisé que dans le cas d'un départ d'un autre médecin. Cette mesure permettrait de renforcer l'accès aux soins dans tous les territoires, en réorientant progressivement les installations des médecins vers les zones intermédiaires

les conditions dans lesquelles les médecins doivent participer à l'accès de tous aux soins, qu'il soit territorial ou financier. La commission a en conséquence émis un avis défavorable sur cet amendement. Quel est l'avis du Gouvernement ? Monsieur

Accepter des patients au-delà de leur patientèle propre, avoir des tarifs maîtrisés ou encore s'engager pour l'accès aux soins non programmés sont des actions menées chaque jour par nombre de médecins dans nos territoires, pour répondre aux enjeux de notre système de santé.

un bon tiers d'entre eux ont déjà ce type d'engagement territorial, cette responsabilité qui fait qu'ils prennent des patients en plus, qu'ils répondent à la permanence des soins, qu'ils s'organisent en cabinet de groupe pour mieux s'organiser et mieux répondre aux besoins de santé de la population.

La commission est évidemment favorable à ce que l'engagement des médecins en faveur de l'accès aux soins soit valorisé. Elle a toutefois jugé ces dispositions à la fois inutiles et malvenues. Inutiles, tout d'abord, parce que la Caisse nationale de l'assurance maladie peut Elle a d'ailleurs commencé à négocier avec les médecins un contrat d'engagement territorial, qui visera à valoriser cette participation sans attendre l'adoption de ces dispositions. ensuite, parce qu'elles interfèrent avec des négociations en cours et aggravent la défiance des médecins. Monsieur le ministre, le jeu de la confiance passera par des négociations apaisées entre la Caisse nationale de l'assurance maladie et les médecins. C'est pour cela, d'ailleurs, que le président Larcher avait demandé que ce texte soit discuté après une négociation conventionnelle. La commission a donc supprimé ces dispositions, qui relèvent largement

Dans le cadre de la lutte contre la covid-19, les préparateurs en pharmacie ont été mobilisés, à titre dérogatoire, pour administrer les vaccins anti-covid, tout d'abord dans les centres de vaccination, puis au sein des officines, sous la supervision d'un pharmacien. Pour favoriser la vaccination contre la covid-19 et contre la grippe saisonnière des personnes pour lesquelles cette double vaccination est recommandée, ils ont également été autorisés à administrer le vaccin antigrippal par l'arrêté du 1 juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Les préparateurs en pharmacie ont donc pu démontrer leur capacité à se former et à vacciner des personnes de tout âge, étant précisé que l'administration des vaccins par les préparateurs en pharmacie formés à la vaccination intervient sous le contrôle effectif d'un pharmacien d'officine.

place pendant la pandémie. Quel est l'avis de la commission ? Les préparateurs en pharmacie ont effectivement été autorisés à vacciner contre la covid-19, la grippe ou la variole du singe à titre dérogatoire, en raison des crises sanitaires, dans les contextes épidémiques que nous connaissons. à titre pérenne cette compétence aux préparateurs en pharmacie. L'administration de ces vaccins par les préparateurs a été très utile depuis 2021, alors que nous menions des campagnes tout à fait volontaristes de vaccination.

la nécessité que cette extension aux préparateurs en pharmacie ne concerne pas les enfants. En effet, cela me gêne un peu que le préparateur en pharmacie puisse vacciner les enfants, qui de ce fait

Le protocole d'accord du Ségur de la santé, plus particulièrement l'accord relatif à la fonction publique hospitalière signé le 13 juillet 2020, prévoit le de la formation des diététiciens, qui nécessite de procéder à la refonte des diplômes. En raison de l'importance croissante de la diététique pour la prévention et la santé de nos concitoyens, les missions des diététiciens sont amenées à se développer. Le besoin d'évolution de cette formation a été rappelé dans un rapport du Haut Conseil de la santé publique en 2017 et dans le programme national nutrition santé (PNNS), qui souligne le nécessaire renforcement du socle universitaire initial au moyen de la validation de la formation au niveau de la licence. Ce besoin d'évolution a également été repris dans le programme national nutrition santé 2019-2023. Dans cette perspective, la formation des diététiciens a évolué, avec la création récente du bachelor universitaire de technologie (BUT) génie biologique, parcours « diététique et nutrition », dont les premiers étudiants seront diplômés en 2024. l'expérimentation d'une licence professionnelle « métiers de la santé : nutrition, alimentation », menée par l'université de Bretagne occidentale est en cours depuis 2022. Cet amendement vise ainsi à introduire une formulation générique pour désigner le diplôme, certificat ou titre requis pour l'exercice de la profession de diététicien, afin de tenir compte des évolutions en cours sur la formation de ces professionnels, en lien avec l'évolution de leurs missions et de leurs compétences. Quel

le décret mentionne qu'il peut s'agir en réalité de deux formations bac+2, le BTS diététique ou le DUT génie biologique option diététique. La création récente d'un bachelor universitaire de technologie, c'est-à-dire un niveau bac+3, dans la perspective d'une montée en qualification, nécessite de modifier en conséquence les conditions légales. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme Florence Lassarade. Renouveler un traitement n'a rien d'anodin, car cela suppose de réévaluer le besoin thérapeutique du patient. Il convient donc de proposer une durée de renouvellement qui ménage l'opportunité pour le patient de bénéficier d'une consultation médicale.

article, qui porte la durée de cette période à trois mois, est assorti de conditions suffisamment encadrées, tenant notamment à l'information obligatoire du médecin prescripteur. Les trois mois de traitement n'étant pas dispensés en une seule délivrance, il est difficile d'imaginer qu'un patient se présente trois fois de suite pour demander une extension de l'ordonnance dans d'autres circonstances que celles d'un

Martine Berthet. L'article L. 6211-3 du code de la santé publique contraint fortement la réalisation des tests, recueils et traitements de signaux biologiques à visée de dépistage, d'orientation diagnostique ou d'adaptation thérapeutique immédiate. Ces différents tests, recueils et traitements de signaux biologiques ne constituant pas des examens de biologie médicale, ils doivent pouvoir être réalisés par les professionnels de santé ou par des catégories de personnes identifiées, et pour simplifier l'accessibilité des patients à ces tests et renforcer la stratégie de prévention et de dépistage. La crise sanitaire a démontré que la stratégie de dépistage est efficace lorsque le patient peut accéder facilement à un test réalisé par un professionnel de santé ou une personne habilitée. Le patient peut ensuite plus rapidement être orienté

? Cet amendement vise à modifier le régime d'autorisation des professionnels de santé pour la réalisation des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne sont pas considérés comme des examens de biologie médicale. Selon le droit en vigueur, un arrêté doit dresser la liste de tous les tests et actes concernés et déterminer les catégories de personnes autorisées à les réaliser. Le présent amendement tend à modifier le régime d'autorisation de ces tests : la liste ne sera plus définie positivement par le pouvoir réglementaire, mais les professionnels prévus par arrêté auront la compétence de principe pour réaliser l'ensemble de ces tests, recueils et traitements. En revanche, un arrêté pris notamment après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) pourra toujours exclure les actes dont la réalisation par ces professionnels de santé ne serait pas opportune. Tout en maintenant des garanties liées à la formation des professionnels autorisés et aux conditions de réalisation, cet amendement tend à assouplir les contraintes du régime actuel, ce qui est souhaitable pour lever les freins aux efforts de dépistage, comme il était possible de le faire dans le cadre de la crise sanitaire.

proposez de modifier la liste des personnes autorisées à réaliser ces tests rapides d'orientation diagnostique, les fameux Trod. Or le code de la santé publique prévoit déjà que ces tests peuvent être réalisés par des professionnels de santé, mais également « par du personnel par du personnel ayant reçu une formation adaptée et relevant de structures de prévention et associatives ou du service de santé des armées ». Ce champ est suffisamment large pour permettre la mobilisation de personnes qui ne sont pas des professionnels de santé, tout en garantissant

vote. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, force est de constater que cette proposition de loi oppose les médecins aux autres professionnels de santé et interroge beaucoup les élus, notamment des zones rurales, sur la coexistence de pratiques différentes en fonction des territoires. Monsieur le ministre, nous devons dire la vérité aux Français : ce texte ne permettra pas de résoudre les difficultés auxquelles certains de nos concitoyens sont confrontés. La démographie des médecins ne s'améliorera pas à moyen terme. Les professionnels de santé mettront plusieurs années avant de s'approprier les innovations prévues par ce texte. Les IPA ne sont pas suffisamment nombreuses- elles sont 1 700 sur l'ensemble du territoire -et la grande majorité d'entre elles exercent à l'hôpital.

cause, je tiens à saluer le travail de notre collègue Corinne Imbert, qui s'est attachée à améliorer ce texte en respectant tous les professionnels- un exercice d'équilibre. Je pense notamment à la suppression des dispositions relatives à la responsabilité collective des professionnels et à la suppression des communautés professionnelles territoriales de santé parmi les structures autorisant l'accès direct pour les IPA et les kinésithérapeutes.

Personne ne demande plus à voter ? ... Le scrutin est clos.